La délégation de compétence permet de confier l'exercice d'une compétence d'attribution à une collectivité ou un EPCI qui dispose de l'expérience, des moyens, mais également de la volonté de l'exercer par simple voie contractuelle. Ce mode d'exercice de la compétence est plus pérenne et sécurisé que les simples conventions de gestion ou de prestations de services. L'élargissement du champ d'application de l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales de revenir à une intercommunalité librement consentie et, surtout, d'apporter de la souplesse et une forme d'adaptation territoriale.

en retenant une telle position, nous saisissons l'occasion d'envoyer un signal fort à nos territoires. Nous voulons rappeler que les échelons de notre administration locale sont et demeureront des maillons essentiels de notre nation.

Plusieurs chefs de filât ont été octroyés à des collectivités territoriales depuis la révision constitutionnelle de 2003. Toutefois, les contours du rôle d'un chef de file sont encore difficilement identifiables. Le texte constitutionnel indique seulement qu'un chef de file dispose, dans un champ de compétences donné, d'une fonction de coordination de l'action de plusieurs collectivités locales habilitées à agir.

lorsqu'elle est en charge d'un service public déterminé, dont elle a la responsabilité exclusive, ou lorsqu'elle dispose d'une responsabilité de planification fixée par le législateur. D'autre part, toute réglementation nationale ou tout document de planification régional ayant pour effet d'encadrer les responsabilités d'une autorité organisatrice,

Le Gouvernement partage l'objectif de clarifier les compétences des collectivités. De fait, la distinction entre compétence exclusive et compétence partagée permet de définir la ligne de partage. La création

Par ailleurs, la rédaction crée des injonctions au pouvoir réglementaire et au législateur potentiellement inconstitutionnelles, sources de complexité et de rigidification. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

associations régies par la loi de 1901 et dont l'objet consiste à soutenir la création et la reprise d'entreprises.

madame la ministre,

Franck Menonville. Les intercommunalités recourent à l'ingénierie des conseils départementaux pour établir leurs projets en matière de développement économique.

Vous le savez, depuis la fusion des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et la création de la CEA, l'Alsace exerce des compétences spécifiques, notamment pour ce qui concerne la coopération transfrontalière et le tourisme, dont elle est désormais chef de file.

La Collectivité européenne d'Alsace, de par sa proximité avec les différents acteurs, est en capacité de mobiliser un réseau d'acteurs fédérés pour mettre en place des projets communs et possède tous les outils pour être chef de file en matière d'économie de proximité. Elle anime et coordonne déjà la marque Alsace, tandis que nos entreprises sont accompagnées et soutenues par l'agence de développement d'Alsace (Adira) et par Alsace destination tourisme (ADT), deux agences travaillant en étroite collaboration avec la CEA.

à ce que connaissent les citoyens et les acteurs économiques sur le territoire.

Ce n'est pas une thématique, mais une modalité d'action, transfrontalière, à propos d'une thématique particulière.

Drexler. Il s'agit d'un amendement de ma collègue Laurence Muller-Bronn. La loi du 2 août 2019 a reconnu la compétence de la Collectivité européenne d'Alsace (CEA) pour promouvoir l'attractivité touristique de son territoire en France et à l'étranger, sans toutefois lui conférer expressément la possibilité d'accompagner à cette fin les entreprises de l'économie touristique. Le présent amendement vise à compléter le dispositif actuel pour le rendre pleinement opérationnel en reconnaissant explicitement, et à moyens constants, la capacité d'action de la Collectivité européenne d'Alsace dans le champ de l'économie touristique et culturelle. Quel est l'avis de la commission

2015. Pour la première fois, à l'occasion des élections de 2020, son assemblée a été élue au scrutin direct. Après six années d'existence, on peut constater un grand nombre de difficultés et de dysfonctionnements dans cette métropole.

conséquent, certains maires, dans des secteurs essentiels comme les transports ou l'urbanisme, se voient opposer par leur minorité ou leur opposition une quasi-interdiction d'aborder des sujets qui sont éminemment communaux.

proposer que soit évalué le fonctionnement de cette métropole, que soient identifiés les dysfonctionnements profonds et que, le cas échéant, soit formulées un certain nombre de propositions pour y remédier. Quel est l'avis de la commission

inconcevable, si je puis dire, et vous le savez bien, de transformer la métropole de Lyon, qui est une métropole à statut particulier, en un EPCI ordinaire,

L'ensemble des communes de la métropole de Lyon doivent pouvoir continuer d'exister, plutôt que de disparaître progressivement dans cette métropole.

Je constate que sur toutes les travées, à l'exception de nos collègues écologistes, il y a un certain accord, à la fois sur le constat et sur la nécessité d'évaluer le fonctionnement de la métropole. En revanche, attendre jusqu'à

Or nous savons tous, y compris les maires de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, quel que soit leur parti, que nous allons droit dans le mur, en particulier à cause du mode électif

Entre 2015 et 2020, la métropole de Lyon a vécu, en réalité, fonctionnellement, sur la base de ce qui existait avant, à savoir la communauté urbaine de Lyon. Les effets réels du nouveau statut peuvent se mesurer depuis l'élection au suffrage universel direct d'il y a un an.

Cet amendement vise à donner un réel pouvoir à la conférence territoriale des maires. Il est moins ambitieux que l'amendement précédent, mais il est très utile.

tous les maires ne sont plus systématiquement « autour de la table » pour régler les problèmes d'intercommunalité. Mon amendement est assez symbolique, mais le symbole a parfois son importance en politique. Je propose de rebaptiser la conférence métropolitaine en « conférence métropolitaine des communes », afin de souligner le fait que les communes, au travers de leur maire, sont associées à la gouvernance de cette métropole.

Du fait de son organisation singulière, les maires ne disposent pas forcément des réponses à apporter à leurs administrés sur les compétences exercées par la métropole. Or ils n'ont aucun contact direct pour les y aider. Le présent amendement vise à créer une sorte de guichet unique, à la métropole, pour les maires, afin de prendre en compte spécifiquement leurs demandes. Au sein de la métropole, les services et les élus sont cloisonnés

d'importantes difficultés, puisqu'ils s'appliquent à des domaines variés pour lesquels l'intervention des maires et la proximité sont plus efficaces. C'est le cas notamment de la police de la circulation. Quel est l'avis de la commission

Par ailleurs, le produit de leur taxe de séjour est réparti sur l'ensemble du territoire, souvent au profit d'autres communes non touristiques. Face à une concurrence étrangère de plus en plus vive, nous devons permettre aux communes touristiques de garder la maîtrise de leur politique touristique.

dans la mesure où cela reviendrait à donner un avantage à la commune qui aura le plus de résidences secondaires dans la composition du conseil communautaire.

transférant de fait la compétence « promotion du tourisme » au niveau intercommunal. Face aux nombreuses difficultés rencontrées sur le terrain quant à l'application concrète de cette mesure, en 2019, le législateur a permis aux stations classées

qui compte autant de communes en littoral que de communes classées « supports de stations de ski », et pour lesquelles il est très difficile de réaliser cette promotion au niveau intercommunal.

pour présenter l'amendement n° 190 rectifié. Si les EPCI disposent normalement de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme », les communes touristiques membres d'une communauté de communes peuvent demander à retrouver cette compétence. Cependant, cette possibilité n'est pas offerte aux communes membres d'une communauté d'agglomération. présent amendement, proposé par Cyril Pellevat, vise à revenir sur cette dissonance en prévoyant cette même possibilité pour les communes membres d'une agglomération, sur le modèle prévu pour les communautés de communes. L'agglomération conserverait concurremment à la commune touristique la compétence « promotion du tourisme », mais à l'exclusion de la création d'offices de tourisme. je vous remercie Cet amendement a pour objet d'accorder la même possibilité aux communes touristiques situées dans les communautés d'agglomération. Une telle disposition va dans le sens de la simplification du droit. En uniformisant davantage le régime de l'intercommunalité, mais surtout en offrant une plus grande liberté, elle permettra d'assurer une meilleure différenciation de nos territoires. La

promotion du tourisme, dont la création d'offices du tourisme » par une simple délibération du conseil municipal. En revanche, pour toutes les communes non classées stations de tourisme, il est nécessaire de passer par une délibération concordante de l'intercommunalité et des communes membres, une procédure beaucoup plus lourde. Pourtant, certaines communes, bien que non classées stations de tourisme, conservent une identité touristique forte et ont une image de marque rayonnant territorialement, voire internationalement. Il est nécessaire que ces communes puissent choisir librement l'organisation touristique la plus adaptée à leur situation. Aussi cet amendement

je vous remercie n° 815 rectifié. Il paraît nécessaire que les communes touristiques puissent décider de retrouver l'exercice de la compétence « promotion du tourisme » quand elles promeuvent une politique touristique ambitieuse sur leur territoire. Aussi, cet amendement vise à permettre aux communes touristiques comptant une capacité d'hébergement d'au moins

En effet, les spécificités des communes touristiques peuvent nécessiter de conserver un pilotage de la promotion et une gouvernance au plus près des réalités locales. À cela, il faut ajouter un contexte international de plus en plus concurrentiel : il est donc essentiel que lesdites communes préservent leur capacité d'action et d'intervention en matière de promotion touristique.

C'est d'autant plus vrai que, depuis que la compétence a été portée au niveau intercommunal, de nombreux systèmes de gestion de la compétence- société publique

de plusieurs délégations et commissions. Nous avons cependant dénombré quelques imperfections juridiques,

l'ouverture des commerces au niveau local. Certaines d'entre elles, issues de la loi dite « Macron » du 6 août 2015, prévoient tout particulièrement des concertations sur le périmètre de chaque schéma de cohérence territoriale Elles concernent notamment l'impact de l'ouverture dominicale sur les équilibres en termes de flux commerciaux et de répartition des commerces sur le territoire.

la possibilité de défendre la revitalisation des centres-villes et de mettre en place, en accord avec les syndicats professionnels et les syndicats de salariés, une régulation intelligente et pertinente de l'ouverture des commerces le dimanche et les jours fériés. Sinon, madame la ministre, les petites villes de demain seront celles d'hier, si ce

et l'intérêt métropolitain. Les domaines d'application sont nombreux et variés, et peuvent concerner le développement économique dans le cas de zones d'activités transfrontalières, ainsi que le transport et les mobilités

souvent qu'ils ne soient pas informés de la répartition des crédits attribués au titre des conventions interrégionales de massifs. Le présent amendement vise à communiquer aux membres de la commission permanente les décisions prises à l'issue de chaque comité interrégional de programmation. Quel

La commission des lois a modifié le mécanisme de délégation de compétence par l'État à une collectivité territoriale ou à un EPCI à fiscalité propre, en supprimant le décret au profit de la seule convention signée par le préfet. J'y suis défavorable, et propose donc la suppression de cet article. Le mécanisme de délégation de ses propres compétences par l'État, dans les formes prévues par le droit en vigueur, est exigeant mais il fonctionne.

Ces décisions étant structurantes pour l'État et présentant des enjeux juridiques, budgétaires, d'organisation administrative nationale et de politique publique, elles appellent une validation interministérielle qui se matérialise par voie de décret.

qui viennent quémander des compétences ou des délégations de compétences, c'est l'État qui soumet ses propositions. À la logique de la demande on adjoint donc une logique d'offre. qu'une telle mesure donne corps au principe de différenciation, puisque le Gouvernement pourra adapter ses propositions selon la spécificité de chacune des régions ou de chacun des départements.

qui suit le renouvellement des conseils régionaux, le Gouvernement soumette à chaque conseil régional une liste de compétences qu'il propose de lui déléguer. C'est ce que j'appelle de la verticalité

la coordination de la politique de l'emploi doit rester une politique nationale, et même une grande cause nationale, avec une stratégie nationale. Nous sommes inquiets de cette volonté récurrente

vous avez souhaité créer un comité national État-régions qui veillerait à l'harmonisation des actions de l'État et des régions en élargissant le champ d'intervention des comités État-région créés par la loi Maptam

(Feader). Les comités État-région existants se justifient évidemment par l'articulation des rôles entre l'État, lequel négocie l'ensemble des éléments financiers juridiques relatifs à ces fonds auprès de l'Union européenne, et les régions, qui ont la charge de leur exécution. Le Gouvernement n'entend pas créer par la loi une instance de concertation générale dédiée au dialogue entre l'État et les régions.

pourrait entraîner une disparition des départements, qui sont pourtant, nous le savons, un échelon de proximité nécessaire, voire incontournable. Par ailleurs, nous ne voulons pas complexifier davantage le schéma territorial, déjà bouleversé par la réforme des nouvelles grandes régions, par la création de collectivités uniques qui ne seraient pas identifiables par nos concitoyennes et nos concitoyens. D'autant plus que ces super-collectivités nourrissent les volontés régionalistes et la mise en concurrence de territoires qui, au nom de leur identité subjective, revendiquent toujours

été rejeté par référendum. Nous privilégions la stabilité de l'organisation territoriale de notre République, avec pour mot d'ordre l'impératif de proximité et de coopération territoriale au sein d'un territoire national subdivisé de la manière la plus harmonieuse possible, et non en différentes entités à statut particulier. C'est pourquoi nous ne souhaitons pas alléger la procédure visant à créer une collectivité unique.

nos concitoyens. Il ne s'agit nullement de créer un nouveau droit des exceptions, auxquelles nous sommes plutôt opposés. Le principe de différenciation est constitutif de l'esprit de la loi.

Vous le savez, en Loire-Atlantique, 105 000 électeurs, citoyens de ce département, se sont prononcés en faveur d'une consultation sur la question du découpage administratif de leur département et de son lien avec la Bretagne.

commission ? Je ne voudrais pas que mon identité bretonne conduise à interpréter la réponse que je vais faire comme un rejet des habitants de la Loire-Atlantique. Plus sérieusement, ces amendements

Cet amendement présenté par notre collègue Ronan Dantec est un parfait préambule aux différents amendements qui seront présentés à l'article 4 relatif à la participation citoyenne.

à une autre région, il est légitime qu'on puisse laisser la région autoriser les habitants de ce département à se prononcer. Ensuite, il reviendra à la région de décider.

répondre à Mme Cukierman, évitons d'avoir des régions organisées autour d'une simple métropole-centre dans une logique de concurrence entre les métropoles, et essayons d'avoir des régions qui ont des capacités de planification

proposée par les rapporteurs affaiblit considérablement les capacités de saisine et les modalités d'organisation des consultations citoyennes.

En effet, dans les municipalités de petite taille, le seuil proposé d'un dixième des électeurs risque de porter atteinte à la bonne administration de la commune. Par exemple, dans une commune de 200 habitants, seulement 20 électeurs suffiraient à provoquer l'inscription d'un sujet à l'ordre du jour du conseil municipal.

Merci

le droit de pétition sera utilisé de manière outrancière par les citoyens. La démocratie locale, c'est un équilibre cela peut, certes, être utilisé par certaines minorités actives, mais cela fait partie du jeu démocratique et on ne peut pas scinder les différentes catégories d'électeurs selon l'endroit où ils habitent.

cela ? Parce que, pour que la participation citoyenne devienne un outil démocratique influent, il faut la considérer comme un outil de gouvernance effectif, à articuler avec le pouvoir politique local.

ce dernier amendement à l'article 4, que le maire informe ses citoyens des modalités pratiques de leur possible participation aux opérations de consultation et pétitions

oubli : l'article 4 du projet de loi abaisse les seuils autorisant les citoyens à solliciter l'organisation d'une consultation au sein d'une commune sans prévoir un dispositif équivalent pour les intercommunalités. Par parallélisme des formes avec l'article 4, nous proposons donc d'assouplir les conditions dans lesquelles les électeurs peuvent solliciter l'organisation d'une consultation populaire au sein des EPCI. Le seuil est actuellement d'un cinquième des électeurs inscrits. Nous proposons de l'aligner sur celui des communes, à savoir un dixième. Nous aurions aimé aller plus loin nous avions initialement proposé de nous aligner sur les nouveaux seuils prévus pour les départements et les régions. Toutefois, après avoir échangé avec la commission, nous avons ajusté notre amendement à 10 % des électeurs. Il s'agit d'un compromis acceptable, qui nous permet d'avancer dans le sens d'une meilleure participation des citoyens à la vie de l'intercommunalité.

tout transfert de compétence des communes vers des EPCI fasse l'objet d'une information du public et d'une concertation dont les modalités sont déterminées par l'assemblée délibérante de l'établissement.

sur la nécessité de passer d'une démocratie à éclipses à une démocratie continue, ce qu'on appelle un processus d'« empouvoirement » des citoyens.

permettant à la fois d'articuler démocratie représentative et démocratie participative et d'ouvrir davantage au public les espaces institutionnels de démocratie locale, qui ne suscitent pas toujours un grand intérêt. Nous constatons tous que la fréquentation,

un maire, avec son conseil municipal, mais pas en assemblée délibérante, d'organiser des réunions publiques et des séances de débat. Cela se fait d'ailleurs non plus en séance, mais dans

il ne s'agit pas d'imposer à chaque citoyen de venir une fois par an devant le conseil municipal pour poser sa question. Il s'agit de faire en sorte que, une fois par an, le conseil municipal puisse accueillir les citoyens qui le souhaiteraient, puissent poser une question orale. Je veux bien que toutes les propositions que nous faisons en matière de démocratie participative soient balayées d'un revers de main ... Mais non ! ... et que, depuis la nuit des temps, nous fassions, les uns et les autres, tout parfaitement dans nos communes. Toutefois, nous avons tous constaté le résultat des élections départementales et régionales, avec la participation la plus faible depuis des dizaines d'années. Nous observons, séquence électorale après séquence électorale, un désamour de nos concitoyens pour la vie publique. Si l'on continue comme ça, on peut fermer la porte

pour renouer le lien entre la démocratie représentative, que nous ne contestons en aucune façon, et nos citoyens, qui ont le droit à la parole dès lors qu'on les autorise à la prendre et que l'on organise des situations dans lesquelles ils puissent le faire.

Je ne sais pas si l'on se rend bien compte du décalage qui existe entre les citoyens et les instances élues. Et si nous ne proposons pas d'outils,

communiquent, voire surcommuniquent sur une démocratie participative qui n'est qu'en fait qu'une réunion où l'on informe les citoyens. D'autres en disent beaucoup moins, mais organisent des réunions où ils construisent

menées dans certaines communes. Je ne me suis pas exprimée sur les budgets participatifs, mais, pour avoir mis en place un budget participatif voilà maintenant cinq ans, je puis vous affirmer qu'il n'existe aucune confusion entre la démocratie représentative et la démocratie participative.

pour économiser le moindre coût est le fil rouge des dernières lois décentralisatrices. Nous l'avons vu avec l'intercommunalisation à marche forcée et la création des grandes régions ; nous le voyons avec le processus de fusion des communes lancé par la loi du 16 décembre 2010 de réforme des La loi prévoit que la création de communes nouvelles dépend uniquement de la décision prise à la majorité dans chacun des conseils municipaux concernés. Un référendum est possible seulement si ces délibérations ne sont pas concordantes. Par cet amendement, nous proposons donc de conditionner la création d'une commune nouvelle à la tenue d'un référendum local, pour que le projet ne se fasse pas contre les habitants des communes concernées par cette fusion, Toujours dans notre volonté de développer la démocratie locale, nous estimons que l'organisation d'un référendum local sur un sujet aussi important doit faire l'objet d'une consultation auprès des administrés des communes soumises à la fusion.

ailleurs, à l'heure où le mouvement de métropolisation fragilise les communes et leurs pouvoirs, il est important de renouer avec une plus grande proximité. Comme pour la création des différents types d'EPCI, si commune nouvelle il y a,

en mettant le citoyen au centre de la prise d'une décision le concernant directement. L'amendement a ainsi pour objet que toutes les communes concernées par la création d'une commune nouvelle doivent organiser une consultation citoyenne. L'avis ainsi rendu- un avis simple, et non conforme -, permettra à l'assemblée délibérante de connaître l'opinion des administrés, sans que cela remette en cause son pouvoir décisionnel. L'association de la population à de tels projets ne ferait qu'en renforcer la légitimité.

avant l'engagement des démarches. C'est la raison pour laquelle nous proposons de mettre en place la possibilité d'une telle consultation, afin de permettre aux assemblées délibérantes des communes de connaître l'opinion des habitants des communes impliquées avant de délibérer.

tout comme dans les autres amendements que nous avons présentés, pourraient faire le choix d'expliquer leurs intentions et de les soumettre à l'avis de la population. La parole est à M. Patrice

particulièrement important pour les citoyens, à savoir la création d'une commune nouvelle, qui interpelle sur l'identité de sa commune. Cet amendement tend à prévoir un avis simple. Bien évidemment, le conseil municipal sera souverainement décisionnaire. Il faut entendre le fait que les citoyens ont envie de participer, surtout sur un sujet comme celui-ci. Malheureusement, très souvent, les citoyens découvrent du jour au lendemain qu'ils font partie d'une commune nouvelle.

commission ? Tout d'abord, nul ne nie ici la réalité de la consultation et de la concertation ! Pour avoir fait un rapport sur les communes nouvelles et avoir traversé toute la France,

telle évolution. La commune nouvelle a cette particularité extrêmement originale d'être une création de l'Association des maires de France, à laquelle, je le souligne, Jacqueline Gourault a largement participé. a largement participé. Nous sommes profondément attachés au fait communal, qui est celui de la proximité et de l'efficacité. Toutefois, il arrive que les communes

avant de prendre des décisions et de délibérer, de consulter la population. Libre au maire de le faire. C'est possible, et même cela se fait

il me semble, pour ma part, que rendre une consultation obligatoire, ou facultative lorsque tous les conseils municipaux ont donné leur accord, malgré l'unanimité, c'est alourdir la procédure. Il vaut mieux stabiliser la situation actuelle.

les conseils de quartier ont fait la preuve de leur utilité. Or, en cette période de défiance démocratique, renforcer la participation est indispensable. Le présent amendement a donc pour objet d'abaisser à 50 000 habitants le seuil

commission ? Vous savez bien que nous n'aimons pas les seuils. Toutefois, les municipalités de moins de 80 000 habitants peuvent créer des conseils de quartier si elles le souhaitent. Nous pouvons donc considérer que l'amendement est satisfait.

biais d'une résolution, saisir le conseil de la métropole pour toute affaire relevant des compétences de celle-ci. Cette faculté ne serait pas limitée à certaines compétences, comme c'est le cas actuellement pour les avis qu'elle rend,

l'installation du conseil régional. Si l'on constate des dysfonctionnements, si la règle n'est pas respectée, c'est un autre sujet, monsieur Lurel. Et vous pouvez, le cas échéant, m'adresser un courrier ; je vérifierai que les choses sont faites comme la loi l'exige. Ce n'est pas par entêtement, mais je persiste et je signe. Je ne conteste pas la liberté de décider d'un règlement intérieur.

ou loi NOTRe, créée en lieu et place de la conférence de coordination des collectivités territoriales par le décret n° 2017-1684 du 14 décembre 2017, ainsi que par l'article 34 de l'ordonnance n° 2016-1562 Cette instance de dialogue entre la collectivité de Corse, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes sur les grands enjeux liés au développement local et territorial avait pour mission première de favoriser la coordination dans l'exercice des compétences respectives des collectivités territoriales territoriales et des différentes intercommunalités de l'île en matière d'action publique et de solidarité financière. C'est en vertu de ces objectifs que, dès son installation, les élus de ladite chambre de l'Assemblée de Corse, notamment ceux de sa commission des compétences législatives et réglementaires, ont acté le principe d'en faire évoluer les statuts, afin de donner à cette institution toute légitimité pour représenter efficacement les territoires et maintenir le niveau intercommunal comme base de la représentation des territoires. La représentativité des territoires est une question particulièrement prégnante pour la Corse, dont la singularité recouvre plusieurs espaces aux contraintes et richesses spécifiques : le littoral et l'urbain, le rural et la montagne. La représentativité des intercommunalités y est d'autant plus cruciale et ne saurait souffrir d'une représentation imparfaite. Forte de ce constat, trois années après la mise en place de cette instance, par une décision du 12 avril 2021, la chambre des territoires a décidé de modifier sa composition, notamment afin d'améliorer la représentativité des communes et de mieux refléter l'égalité entre les

le 20 mai 2021.

ce sont vos propres mots. Alors que la collectivité de Corse vous propose que ce lieu soit la chambre des territoires, vous refusez ! J'ai du mal à le comprendre ...

1688. Le présent amendement vise à renforcer

un dispositif très précis, avec étude d'impact et, ils ne seraient pas en mesure de prendre une délibération en toute connaissance de cause. Bien sûr ! S'ils prennent des délibérations concordantes, c'est évidemment qu'ils en auront étudié les impacts et qu'ils en auront fait le choix. Pourquoi un

Je serai bref, car M. Pointereau a dit l'essentiel. Que des gens ne soient pas condamnés sans cesse à travailler ensemble alors qu'ils ne le veulent plus

Il ne faut pas croire, chers collègues, que c'est uniquement parce que deux personnes seraient en conflit qu'il y aurait des demandes de scission. Il appartient au préfet et aux élus de conduire une réflexion. Je rappelle que ce n'est le fait ni d'un président d'EPCI ni d'un maire, puisque des délibérations doivent être prises au sein de l'EPCI et des communes et qu'elles doivent être concordantes sur des périmètres.

et les études d'impact- cela a été dit -sont prévues. Tout a été fait dans les règles. Or on a tout de même le sentiment, madame la ministre, et vous ne m'enlèverez pas cela de la tête- j'ai des exemples factuels sur d'autres sujets, comme la subdélégation -, que tout est fait parfois par les services de l'État pour décourager les élus Je m'empresse de dire à mon collègue Éric Kerrouche que, s'il y a des divorces qui coûtent cher, il y a aussi des mariages, à la suite de la loi NOTRe, qui ont coûté très cher, parce que les études d'impact ont été passées sous le tapis

rectifié . Le présent amendement, proposé par notre collègue Fabien Genet, vise à renforcer l'intérêt de la conférence des maires, en prévoyant les cas dans lesquels cet organe doit être consulté pour avis, préalablement à l'adoption d'une délibération par l'organe délibérant. Ces cas concernent les grandes décisions stratégiques de l'intercommunalité pour lesquelles les maires des communes membres doivent être entendus.

de prévoir la liste des cas dans lesquels la conférence des maires doit être consultée, mais que c'est à l'intercommunalité de le faire en début de mandat. À titre d'exemple, le conseil communautaire pourra décider que la conférence des maires devra être consultée avant l'adoption de toute délibération relative à la modification des statuts de l'EPCI,

de la commission ? Comme M. Marie, je déclare ma foi et ma confiance dans l'intelligence territoriale et la libre administration des territoires, mais je n'arrive pas du tout aux mêmes conclusions que lui

En effet, nous étions conscients que certaines intégrations de communes posaient problème et étaient contraires à une logique de bon sens. Seulement, en voulant simplifier la loi, nous avons intégré un seuil d'habitants minimum

Votre amendement a pour objet de créer un seuil de population de 30 000 habitants pour les communautés d'agglomération dérogatoire à celui qui

ne saurait être autorisé s'il a pour conséquence un passage en dessous des seuils de population, qu'il s'agisse d'un retrait de droit commun ou d'un retrait dérogatoire. Il n'apparaît donc pas opportun de créer

cela affaiblirait les fondements des communautés d'agglomération, dont l'importance de la population est l'un des critères justifiant leurs compétences plus intégrées que celle des communautés de communes. Le Gouvernement

de notre collègue Kerrouche, cette proposition ne nous paraît pas souhaitable, d'autant que les régions sont déjà libres d'organiser un référendum local.

l'initiative de la collectivité dont les modalités relèvent de la loi organique. Le dispositif proposé relève donc, à mon sens, de la loi organique et non de la loi.

: La parole est à M. Hervé Marseille. Les délégués élus par les conseils municipaux dans les organes délibérants des syndicats de communes sont désignés suivant les modalités prévues par l'élection du maire. Cette disposition est adaptée lorsqu'il n'y a qu'un unique délégué titulaire au sein de l'organe délibérant. En revanche, elle est particulièrement complexe à mettre en oeuvre lorsque l'organe délibérant comprend de multiples représentants de chaque membre.

syndicats. Pour la composition du comité syndical, il tend à appliquer les mêmes règles que celles qui sont prévues pour la représentation des communes dans les organes délibérants des communautés de communes et des communautés d'agglomération, par renvoi aux dispositions de l'article L. 5211-6-1 applicables à la répartition des sièges des conseillers communautaires. je vous remercie

Dans un souci de simplification et par cohérence, le présent amendement a pour objet que la représentation-substitution d'une communauté à ses communes membres au sein d'un syndicat mixte oeuvrant dans des domaines de compétence qu'elle exerce devienne une conséquence mécanique de ses évolutions statutaires. Je le répète, cette disposition est une mesure de simplification.

des dispositifs de démocratie directe. À l'heure où la crise de confiance à l'égard des élus et la désaffection des citoyens pour les urnes n'ont jamais été aussi grandes, nous devons autoriser les collectivités qui le souhaitent à développer des instruments de démocratie locale.

Le droit à l'expérimentation découle de la révision constitutionnelle de 2003 : il permet aux collectivités de déroger aux lois et règlements dans des conditions strictes et très encadrées. Seules quatre expérimentations ont été conduites depuis cette date, dont trois ont été généralisées : le revenu de solidarité active, la tarification sociale de l'eau et l'accès à l'apprentissage jusqu'à l'âge de 30 ans.

Pour poursuivre nos efforts dans ce sens, il est proposé d'inscrire les dispositifs de démocratie directe dans le champ des expérimentations que peuvent mener les collectivités locales. Quel l'avis de la commission ? Je comprends l'attachement de nos collègues à la démocratie directe. Toutefois, il nous semble à ce stade que de nombreux outils, comme le référendum local,

suggérait des modalités d'entrée et de maintien dans l'emploi qui sont totalement étrangères à la réalité du mandat politique. Cette réflexion a déjà fait l'objet de débats à l'occasion de la loi Engagement et proximité. Par conséquent, j'émets un avis défavorable

En faisant passer le nombre de régions métropolitaines de vingt-deux à treize, cette loi a vraisemblablement accentué le désintérêt des Français pour l'échelon régional. lors, est-il surprenant qu'un texte ayant créé une strate territoriale aussi étendue que floue et fusionné une myriade de services, au détriment d'une logique de proximité, ait de telles répercussions ?

Cet article permet un transfert « à la carte » de compétences supplémentaires à un établissement public de coopération intercommunale par les communes J'y suis défavorable, car cet article conduirait à revenir en arrière et à annuler près de cinquante ans d'intégration et de mutualisation des compétences, ainsi que de renforcement de la solidarité dans le cadre de l'intercommunalité. En effet, les intercommunalités ne pourraient pas fonctionner de manière efficace dans le cadre qu'instaure cet article. Tout d'abord, cette situation serait peu lisible. lisible. Les citoyens, même ceux qui habitent dans des communes voisines, ne voteraient pas pour les mêmes enjeux aux élections municipales. Ensuite, la gouvernance deviendrait difficilement gérable, puisque les élus ne voteraient pas sur l'ensemble des sujets. Enfin, sur un plan financier, le calcul des compensations serait extrêmement complexe.

Pour autant, chacun des conseillers communautaires élus au suffrage universel se prononce ensuite sur l'ensemble des missions et des compétences exercées par l'EPCI. De nombreux autres mécanismes, comme la définition de l'intérêt communautaire ou les dispositifs de mutualisation, concourent également à cette flexibilité que nous appelons toujours de nos voeux. Dès lors, il ne me paraît pas souhaitable de mettre en oeuvre un transfert de compétences à la carte,

Il est issu des remontées des conférences des maires, que la loi Engagement et proximité a encouragées. L'intercommunalité a atteint un niveau de maturité qui permet aujourd'hui de promouvoir une vision plus moderne et plus souple de l'exercice de ses compétences et des politiques publiques. Afin de mieux prendre en compte les situations locales, cet amendement a pour objet que les intercommunalités qui le souhaitent, souvent des EPCI de grande taille, puissent intervenir dans un domaine de compétence facultatif sur une partie de leur territoire, autant contraindre l'ensemble des communes à opérer un tel transfert de compétences. Il tend à adapter en conséquence les règles de gouvernance ou de financement de ces compétences. Le conseil communautaire définirait une liste des compétences ou parties de compétences susceptibles d'être transférées à la communauté, et chaque conseil municipal pourrait demander, ou non, le transfert de tout ou partie de ces compétences. Le transfert serait ensuite décidé par délibération concordante du conseil communautaire et de l'ensemble des conseils municipaux, selon la règle de la majorité de droit commun.

la France comporte toujours 18 377 communes de moins de 500 habitants et 3 349 communes de moins de 100 habitants. L'atomisation communale est une réalité française. La contrepartie de cette atomisation, c'est la force démocratique

d'activité économique : les rapporteurs souhaitent que l'on en revienne à la situation antérieure, celle d'une concurrence systématique entre communes, avec l'impossibilité de mettre en place des schémas

l'article 4 . Le rétablissement du critère de l'intérêt communautaire ou métropolitain pour la détermination de certaines compétences transférées aux EPCI à fiscalité propre constituerait un retour en arrière majeur et un « détricotage

permettent aujourd'hui de définir des stratégies de développement économique à l'échelon de l'intercommunalité qui seraient remises en cause si l'on en revenait

. Cet amendement vise à clarifier la répartition des compétences entre les communautés de communes et communautés d'agglomération, d'une part, et leurs communes membres, d'autre part, en matière de commerce. Il s'agit de préciser, actuelle, que la politique locale du commerce relève de la compétence de l'intercommunalité, alors que le soutien aux activités commerciales est soumis à la définition d'un intérêt communautaire.

Cet amendement vise à corriger un oubli de la loi NOTRe et à étendre la compétence relative à la politique locale du commerce des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre aux métropoles, afin que celles-ci puissent définir une stratégie métropolitaine en la matière. S'agissant du soutien aux activités commerciales, un intérêt métropolitain doit pouvoir être défini, afin de permettre aux communes de continuer à agir dans ce domaine.

Face à l'échec de la commission de conciliation actuellement prévue par le code de l'urbanisme, la commission des lois, par l'intermédiaire d'un amendement de Rémy Pointereau, a souhaité la remplacer par une conférence de dialogue aux attributions plus larges. Cette nouvelle instance aurait ainsi un pouvoir d'arbitrage. Il s'agirait d'instituer une saisine obligatoire de ladite conférence préalablement aux déférés préfectoraux, avant de saisir le tribunal administratif

est contraire à la Constitution, laquelle confie aux seuls préfets la prérogative d'exercer le contrôle administratif sur les collectivités territoriales et le soin de décider de l'opportunité de déférer les actes qu'ils estiment illégaux. En pratique, le déféré préfectoral intervient toujours comme ultime étape après un désaccord, si je puis dire, entre l'État et les collectivités territoriales. Il est systématiquement précédé d'un dialogue, voire de négociations,

le droit de l'urbanisme organise d'ores et déjà des séquences obligatoires de dialogue entre l'État et les collectivités territoriales. Le dernier exemple en date est l'introduction, dans le droit positif, de la note d'enjeux, exigée dans le cadre de l'élaboration des schémas de cohérence territoriale

Les administrés ne sont malheureusement pas au fait des différentes compétences des collectivités locales composant leur territoire, et ce d'autant plus qu'elles ne sont en rien uniformes et dépendent des décisions des collectivités concernées. Cette méconnaissance contribue malheureusement à éloigner les citoyens des décisions qui les concernent. Aussi, il paraît utile que soit élaboré un document, accessible au grand public, permettant à chaque administré de comprendre les schémas d'élaboration des décisions qui ont un impact sur son quotidien. L'article 4 , introduit en commission, crée une conférence de dialogue entre l'État et les collectivités Nous y voyons une opportunité, dans la perspective de rapprocher les administrés des administrations. Cette conférence pourrait ainsi élaborer, à destination du grand public, un document accessible recensant les compétences de chacune des collectivités territoriales. Tel est le sens de cet amendement. Quel est l'avis de la commission

montagnards, vise à créer un code de la montagne. Celui-ci réunirait, dans un même ouvrage, les différentes dispositions contenues dans les lois, codes et autres textes réglementaires qui concernent les territoires de montagne, afin de les rendre visibles et accessibles à tous. législateur a exprimé cette volonté à l'article 79 de la loi du 5 janvier 2006 d'orientation agricole dans les termes suivants : « Les dispositions législatives et règlementaires relatives au domaine de la montagne sont regroupées dans un code de la montagne. Face à l'inertie des services de l'État, qui n'ont pas rédigé le code de la montagne attendu par les montagnards, l'Association nationale des élus de la montagne a réalisé en 2014 un « code éditeur », avec la caution de la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique. Aujourd'hui, plus de quinze ans après la publication de la loi, il faut la respecter dans toute sa rigueur en rassemblant

de vote. Je regrette que l'on n'ait pas eu de mots assez gentils pour vanter les vertus de la proximité et de l'efficacité. Cet amendement vise simplement à ne pas imposer une irréversibilité : ce qui est vrai à une époque